J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Marcel Rainaud, qui fut sénateur de l'Aude de 2006 à 2014. J'ai le souvenir du fauteuil qu'il occupait, après avoir succédé à Raymond Courrière. J'ai aussi le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Christian Bonnet, qui fut sénateur du Morbihan de 1983 à 2001. J'évoquerai sa mémoire dans quelque temps. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mardi 21 avril, après-midi et soir, sous réserve de son dépôt et de sa transmission, du projet de loi de finances rectificative pour 2020 et, à l'ordre du jour du jeudi 23 avril, matin, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020 ou l'examen en nouvelle lecture de ce projet de loi. Acte est donné de ces demandes. Le délai limite pour le dépôt des amendements de séance en première lecture serait fixé au mardi 21 avril à l'ouverture de la discussion générale. La durée de la discussion générale pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire ou la nouvelle lecture pourrait être fixée à quarante-cinq minutes. En cas de nouvelle lecture, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance serait fixé au jeudi 23 avril à l'ouverture de la discussion générale. Y a-t-il des observations ?

Comme à l'habitude, nos collectivités sont au rendez-vous. Elles produisent un effort inédit, serein, mais déterminé, rigoureux et résolument tourné vers le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles et les plus démunis. Elles se préoccupent aussi grandement du tissu économique de leur bassin de vie. Car, si la lutte sanitaire est la priorité, la reprise de l'activité économique est le second pilier qui doit guider la reconstruction. Notre économie devra tirer toutes les leçons de nos échecs passés et des impensés d'une mondialisation béate, pour devenir enfin plus respectueuse de notre environnement et résiliente. Ce mot résonne pour moi particulièrement dans cet hémicycle aujourd'hui, puisque mon groupe

Fonds de soutien métropolitain d'urgence aux entreprises et à l'emploi, comme à Bordeaux, exonération du paiement de la redevance d'occupation du domaine public ou de loyers communaux dans des centaines de mairies, fonds de la région Occitanie et de tant d'autres : les collectivités se surpassent face à la crise, car, sans leurs interventions, c'est l'entièreté de notre écosystème qui sombrera. Les élus locaux savent mieux que quiconque quelle politique publique mener en proximité, dans cette République des territoires si chère aux radicaux et au président Gérard Larcher, qui a évoqué si justement ces « petites Républiques dans la grande Alors, aux fins de donner durablement corps aux annonces du Président de la République, ainsi qu'à l'esprit du projet de loi 3D- décentralisation, différenciation et déconcentration -, qu'il envisageait de présenter avant l'état d'urgence, quels moyens et quelles compétences le Gouvernement entend-il donner à la France des collectivités ?

nous avons d'abord permis aux collectivités d'exécuter leur budget dans des conditions beaucoup plus souples qu'habituellement, comme l'avait d'ailleurs demandé le Sénat lors de l'examen du projet de loi d'urgence Pour mémoire, je citerai la possibilité d'exécuter des dépenses de fonctionnement comme d'investissement avant le vote du budget, reporté, comme vous le savez, à la fin du mois de juillet ; le pouvoir confié directement à l'exécutif local de souscrire des lignes de trésorerie ou d'attribuer des subventions aux associations, qui jouent aussi sur le terrain un rôle très important ; et le pouvoir donné aux présidents de région d'attribuer directement des aides aux entreprises. Par ailleurs, le Gouvernement a immédiatement pris la décision de suspendre les contrats dits de Cahors de maîtrise de la dépense publique, conscient de la pression qui risque d'être exercée sur les dépenses de fonctionnement des collectivités En outre, des mesures ont été prises dans le champ des aides aux entreprises. Vous le savez, un fonds national de solidarité a été créé, financé principalement par l'État à hauteur de 5,5 milliards d'euros, mais aussi par les régions, pour un montant de 500 millions d'euros. Une dérogation ponctuelle et exceptionnelle à la répartition des compétences des collectivités en matière d'aide aux entreprises permet aux communes, aux EPCI et aux départements de participer au fonds par convention avec l'État. Enfin, État et collectivités doivent s'organiser pour que les entreprises disposent d'interlocuteurs bien identifiés, dans une logique de guichet unique. Je veillerai bien sûr à l'avenir à ce que les collectivités qui participent soient dûment associées aux procédures et informées des aides accordées sur leur territoire. ce n'est que dans une logique partenariale très forte qu'État et collectivités trouveront les solutions les plus adaptées pour préparer l'avenir de nos territoires. Le Gouvernement veut ainsi répondre à la crise qui nous touche, pour nous préparer à

et de la jeunesse, depuis le début de l'épidémie, les décisions du Gouvernement s'appuient sur l'expertise de scientifiques. Pouvez-vous nous communiquer l'avis scientifique indiquant la pertinence d'une réouverture des établissements scolaires le 11 mai prochain ? Pouvez-vous nous dire quels seront les enfants prioritairement invités à aller à l'école, puisque vous avez indiqué que cette reprise ne serait ni simultanée ni obligatoire ? Pouvez-vous nous dire quels matériels et quelle quantité de matériels seront mis à disposition des personnels de l'éducation nationale comme des agents territoriaux ? Les soignants manquent encore de tout aujourd'hui, ce qui est très inquiétant. Quelles consignes et quels moyens seront donnés aux collectivités pour assurer l'entretien ou la désinfection régulière des locaux ? Devront-elles assurer la restauration ou le transport scolaire ? en matière de test ? Il semble que les enfants et les jeunes soient porteurs asymptomatiques du Covid-19. Si l'on veut enrayer l'épidémie, il paraît donc indispensable de les dépister, tout comme le personnel enseignant. Tout semble indiquer, monsieur le ministre, que la date du 11 mai

proposé, les fermetures de classes dans les zones d'éducation prioritaire à la prochaine rentrée. Il faut doter nos collèges et lycées de postes supplémentaires, alors que certains sont supprimés. Voilà comment on résoudra les inégalités sociales dans l'école ! Je crains que les Français qui pensent aujourd'hui

exacerbe les inégalités ; comme toutes les crises, en effet, elle frappe d'abord et surtout les plus fragiles, les moins protégés. Des femmes et des hommes sont aujourd'hui abandonnés à leur sort. Je pense aux sans domicile fixe, aux migrants, aux populations roms, qui vivent dehors, dans des squats, des bidonvilles ou des campements de fortune, mais aussi dans des centres de rétention. Alors que le confinement et la distanciation sociale sont nos principales armes contre l'épidémie, ces mesures sont inapplicables dans ces endroits, où les conditions de vie et d'hygiène sont désastreuses. Une centaine d'associations et d'ONG (organisations a saisi les Nations unies pour demander au gouvernement français de mieux inclure ces personnes dans la gestion du coronavirus. Je pense aussi à ces autres invisibles que sont les familles monoparentales, les étudiants et les jeunes, qui ne bénéficient pas du RSA en fin de droits et précaires, souvent exclues du numérique. Les maires et les associations font un travail exceptionnel pour répondre à ces problématiques, mais les moyens sont insuffisants. Dix-neuf présidents socialistes de département ont réclamé l'instauration d'un revenu de base universel pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté et amortir le choc social prévisible. Le Gouvernement a mis beaucoup d'argent sur la table pour éviter le naufrage économique, alors même que les actionnaires continuent de percevoir des dividendes. Mais il doit aussi éviter le naufrage social. Déjà un mois de confinement, et les invisibles que j'ai évoqués n'ont eu droit qu'à bien peu d'égards. Vous venez juste de décider une aide exceptionnelle qui ne peut rien résoudre dans la durée et ne concerne que les familles avec enfants. Pourtant, une société se grandit quand elle prend soin des plus fragiles.

ce sont près de 10 000- je dis bien 10 000 -places d'hôtel que nous avons réquisitionnées. Hier soir, 174 000 personnes ont été accueillies et mises à l'abri dans les centres d'hébergement d'urgence. Pour celles et ceux qui sont atteints du Covid-19 mais qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, nous avons créé, avec les associations, que je salue, plus de 80 sites partout sur le territoire, en métropole et dans les outre-mer.

Beaucoup de Français veulent déjà être prêts pour l'après. Qu'ils soient en première, en deuxième ou en troisième ligne, la pandémie n'a pas entamé leur volonté de construire le futur. Je salue ici leurs efforts et leur discipline. Nous leur devons un langage de clarté. Cela vaut notamment pour le bâtiment. Le secteur est particulièrement affecté par la crise qui paralyse notre économie. Pour de très nombreuses entreprises, le coup d'arrêt est brutal. Même si les chantiers reprennent au cas par cas, lorsque les conditions sanitaires sont réunies, de nombreux patrons craignent pour leurs employés et pour la survie de leur entreprise. Outre ces difficultés actuelles, des préoccupations surgissent déjà concernant l'avenir et la reprise future des activités. En effet, à la suite de la neutralisation des délais administratifs, de nombreuses collectivités territoriales ont suspendu l'instruction des dossiers de permis de construire. Sachant que les délais de recours demeureront incompressibles, les retards qui s'accumulent aujourd'hui devront être purgés le moment venu. En outre, la prorogation d'un mois des délais d'autorisation après la fin de l'état d'urgence sanitaire risque d'aggraver la donne. Monsieur le ministre, que compte faire le Gouvernement pour éviter un faux départ au moment du déconfinement ? La situation est trop grave pour que nous nous permettions d'ajouter aux difficultés actuelles des difficultés futures.

Je m'interroge et je vous interroge, monsieur le Premier ministre, sur la stratégie française qui consiste à tout miser sur le confinement. Entendez-moi bien ; la stratégie du confinement est indispensable, notamment pour soulager nos hôpitaux, mais elle a d'énormes effets collatéraux.

je vous le demande : à partir de quand notre pays, la France, pourra-t-il enfin combiner une stratégie défensive avec une stratégie offensive ? C'est ce que font les pays qui ont eu du succès.

d'une pression considérable et d'efforts absolument admirables, mais il a tenu. Cela dit, nous ne nous sommes pas cantonnés à organiser le confinement et à attendre, ensuite, que les choses se passent, vous l'imaginez bien.

de début mai jusqu'à fin juin, selon des modalités totalement inédites, des modalités que nous sommes en train, en quelque sorte, d'inventer ; ce ne sera pas la classe comme avant. Cela permet de répondre à une bonne partie de vos questions. D'abord, pour

essentiel. Mais d'ores et déjà, et ils le démontrent dans la crise, nos institutions et nos agents publics sont aujourd'hui en première ligne pour assurer la continuité des services essentiels à notre nation. Au-delà, ils maintiennent l'unité du pays, ils le tiennent debout, ils garantissent l'attention à chacun, la concorde et la paix. Le Président de la République confiait au Gouvernement des décisions dans des délais rapides, notamment pour soutenir plus avant le secteur privé, particulièrement les libéraux et les indépendants,

aux enseignants, qui maintiennent un lien essentiel là où les inégalités sociales sont les plus fortes et les plus criantes en ce moment. Nous pensons aussi aux très nombreux fonctionnaires, notamment d'État et territoriaux, que l'on cite moins. Ils prennent des risques. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils font souvent face à une surcharge de travail importante, notamment les services sociaux, la protection de l'enfance, la justice, les centrales ministérielles, les fonctions support, la collecte d'ordures ménagères, les CCAS

une prime exceptionnelle existe pour les salariés du privé. Une prime pour les agents publics des trois versants est annoncée. Elle est légitime. Elle est attendue. Pouvez-vous nous en préciser les critères d'attribution, les modulations et les délais de mise en oeuvre ? La parole est à M.

chacun des exemples que vous avez cités témoigne de l'importance de l'action des agents publics titulaires et contractuels dans notre quotidien, pour assurer la continuité de la vie de la Nation. Votre question est l'occasion pour moi de les en remercier

Le Président de la République avait indiqué sa volonté de reconnaître l'engagement des agents dans cette période de crise, notamment pour celles et ceux qui font face à un surcroît d'activité. Sous l'autorité du Premier ministre, nous avons travaillé en ce sens. Les fonctionnaires hospitaliers, les personnels soignants et non soignants bénéficieront du paiement rapide et majoré des heures supplémentaires, comme l'a souligné le ministre des solidarités et de la santé. Ils bénéficieront également du versement d'une prime plus forte dans les territoires et les hôpitaux particulièrement confrontés au virus du Covid-19, mais aussi dans l'ensemble des territoires.

Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, à la demande de très nombreuses associations d'élus, nous avons créé la même possibilité : une prime défiscalisée et désocialisée, d'un montant maximal de 1 000 euros,

C'est une reconnaissance matérielle de l'engagement des agents, qui s'ajoute à la reconnaissance et à l'hommage moral que nous leur rendons les uns et les autres. L'engagement est ainsi tenu

On ne peut malheureusement que souscrire à son propos tant les failles et les insuffisances sont nombreuses. Elles vont bien au-delà de notre système de santé. La crise s'est comportée comme un révélateur et les difficultés que rencontrent les personnes les plus fragiles nous ont sauté aux yeux. La situation dans les Ehpad a témoigné de notre très grande difficulté à protéger nos aînés. La crise a montré de façon criante l'écueil que constitue pour la personne handicapée l'accès aux soins. Ce n'est pas simple en temps normal ; c'est devenu presque impossible en temps de crise. La fermeture des internats pour enfants en situation de handicap a conduit au retour d'enfants au domicile de leurs parents, entraînant pour ces derniers une situation délicate. Là encore, la crise a mis le doigt sur le manque de moyens d'accompagnement que connaissent trop souvent les proches aidants. Nous pourrions également évoquer les difficultés grandissantes des Français les plus pauvres, des mères isolées, des travailleurs précaires, des mal-logés Monsieur le ministre, si le confinement n'est pas toujours facile à vivre pour les Français, il l'est encore moins pour les plus fragiles d'entre eux. De ce point de vue, la pandémie aura joué un rôle de révélateur implacable. Quelles leçons vis-à-vis des plus fragiles comptez-vous tirer Dans son allocution, le Président de la République a vanté, ce qui est nouveau, les vertus du port du masque pour tous. Dont acte ! Il a indiqué que les masques seront distribués par les communes, mais il n'a pas été précis sur certains points. D'où viendront ces masques ? Qui les financera ? Les maires se posent déjà des questions. Certaines communes ont pris les devants et ont commencé à acheter des masques, en priorité pour le personnel médical. Ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable qu'elles bénéficient pour ces achats d'un taux de TVA réduit ? Enfin, monsieur le ministre, nous avons bien compris que le confinement est pour l'instant la seule véritable réponse que nous sommes en mesure d'opposer à la maladie. Cela met en grande difficulté les professionnels du tourisme.

de solidarité à destination des 4 millions de foyers les plus précaires de notre pays. Sont concernées les familles avec enfants, mais aussi les travailleurs pauvres et les bénéficiaires du RSA. Tous les bénéficiaires du RSA et de l'ASS percevront 150 euros de prime,

L'inquiétude est forte ; mes collègues s'en sont fait l'écho à travers leurs questions. Le sentiment qui domine aujourd'hui est encore celui de l'impréparation du Gouvernement. Vous renvoyez la définition des conditions précises requises pour préserver la santé des enfants et des personnels à la concertation.

Peut-on demander à des enfants de maternelle de respecter les gestes barrières ? Peut-on demander à un enseignant d'apprendre à écrire à un enfant en restant à un mètre de lui ? Pourquoi envisagez-vous de rouvrir les écoles primaires avant les collèges et les lycées ?

global, général, très ambitieux à la rentrée scolaire pour lutter véritablement contre les inégalités sur le long terme. Ce n'est pas à quelques semaines du mois de juillet que l'on résoudra les problèmes posés par le confinement.

pour que la crise sanitaire ne nous fasse pas passer d'une société de la bienveillance à une société de la surveillance, pour que le recours au numérique dans la sortie de crise soit efficace, il faut créer de la confiance avec les Français. Pour atteindre cet objectif, la mise en place d'une application, sur mobile, de traçage des contacts sociaux ne peut donc se faire dans notre pays que sur la base de trois éléments cumulatifs. Premièrement, la préservation des libertés. En prononçant les mots « volontariat » et « anonymisation », le Président de la République a donc confirmé que cette solution se ferait dans le cadre du respect aussi bien du droit national que du droit européen, notamment du RGPD Deuxièmement, la recherche de l'universalité. Pour être efficace, cette application ne doit pas concerner uniquement les personnes familières des nouvelles technologies. seulement faire preuve de pédagogie pour rassurer nos concitoyens et les inciter à utiliser cet outil, mais aussi se préoccuper dès maintenant des moyens humains qui devront accompagner le déploiement de ce dernier. Corée, pas moins de 20 000 personnes ont mené ce travail. Se reposer uniquement sur le numérique n'aurait pas de sens, notamment parce qu'il faudra aussi alerter des personnes qui n'auront pas recours à cette application Troisièmement, la protection de notre souveraineté. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans cette crise du Covid-19, mais nous disposons, par exemple avec nos amis allemands et suisses, de toutes les compétences pour que la solution informatique soit française et européenne. Sur ce dernier point, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous confirmer que l'intégralité de l'infrastructure informatique sera sous notre propre contrôle- l'application elle-même, l'hébergement des données ou le capital des entreprises chargées de sa réalisation ? En d'autres termes, sommes-nous capables et avons-nous la volonté de résister aux assauts des géants du numérique pour offrir aux citoyens français une réponse nationale dans laquelle ils pourront avoir vraiment confiance ? La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du numérique.